Monsieur le président, La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales, présentée par Mme Nathalie Delattre, M. François Pillet et plusieurs de leurs collègues Dans la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Delattre, auteure de la proposition de loi. Monsieur

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que de chemin parcouru ! Que de travail accompli depuis la rédaction de cette proposition de loi déposée le 30 juillet 2018, voilà presque un an,

avait accepté de me parrainer et de me conseiller dans le cheminement de ce texte de loi, un appel cosigné par près de 20 % d'entre nous. Nous avions alors pour objectif de porter au coeur de cet hémicycle le débat sur le rôle que peut jouer la médiation territoriale, aux fins de rapprocher l'administration de ses administrés. Entre-temps, cette proposition de loi a rencontré l'actualité. Elle a trouvé un écho particulier à l'échelle nationale, avec le mouvement des « gilets jaunes ». Cet élan de protestation a mis en lumière, sur l'ensemble de notre territoire, l'extrême défiance de nos concitoyens envers nos mécanismes démocratiques.

a répondu de manière originale à cette crise, en organisant un grand débat national. Ce sont près de 700 médiateurs, 700 facilitateurs de parole, qui ont eu la lourde tâche de transformer une contestation violente en une concertation constructive. Ce sont eux qui ont eu la responsabilité d'animer et de réguler au plus près du terrain ces participations de citoyens aspirant à devenir bien plus que de simples administrés- la responsabilité de redonner de la vitalité à notre démocratie. C'est pourquoi, dans le cadre du grand débat national organisé au Sénat, j'avais tenu à interroger Mme la ministre de la justice, Nicole Belloubet, sur l'opportunité de notre proposition de loi et sur le rôle des médiateurs territoriaux au sein au sein de nos collectivités locales. Dans sa réponse, Mme la garde des sceaux avait reconnu le rôle que pourrait jouer la médiation territoriale, pour « revivifier l'expression de la citoyenneté en France ». La médiation territoriale a d'ores et déjà fait ses preuves sur notre territoire : elle apparaît comme le maillon manquant entre les administrations et leurs résidents. Même s'il est difficile de recenser les médiateurs, car ils ont des statuts et des pratiques pouvant différer, l'Association des médiateurs des collectivités territoriales en dénombre une quarantaine

comment développer au mieux ce formidable outil qu'est la médiation territoriale ? Comment instiller cet élément de réconciliation dans nos rouages administratifs, sans créer une nouvelle charge pour nos collectivités ? C'est tout le travail que nous avons mené avec le rapporteur François Bonhomme, que je salue et remercie chaleureusement de son attrait et de sa réelle implication dans cette cause. C'est aussi le fruit de nombreuses sollicitations que nous avons spontanément reçues à la suite de la publication du texte en juillet 2018. Je souhaitais donc tout naturellement remercier les associations de médiateurs et les représentants d'acteurs de la médiation territoriale que nous avons auditionnés et qui ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est sans oublier l'appui du ministère de la justice et le vif intérêt manifesté par M. le ministre Sébastien Lecornu, qui a tenu à être présent aujourd'hui. Nous n'avons pas eu la prétention d'embrasser l'ensemble des problématiques de la médiation française. L'objectif était de réunir des textes épars et de les enrichir sur le seul champ de la médiation territoriale. Nous avons saisi l'occasion de ce véhicule législatif pour élaborer un socle solide, capable de faire prospérer écoute et dialogue au sein de nos collectivités et de faire naître de nouvelles initiatives de règlement de conflits au quotidien. Cette disposition est attendue, car elle va permettre de limiter le nombre de recours juridiques et de régler certains vices de procédure, parfois chronophages.

Si cette obligation, initialement prévue dans la proposition de loi, pouvait favoriser un développement rapide de ce mode de résolution à l'amiable, nous avons décidé d'éviter toute nouvelle contrainte pour les collectivités territoriales. Ce texte permet de parvenir à une notion de médiation territoriale, dans laquelle le rôle du médiateur y est défini par son champ de compétences. Nous avons pris le parti d'exclure les différends avec les autres personnes publiques et les litiges internes de gestion des ressources humaines. Nous avons également tenu à articuler son action avec celle du Défenseur des droits, dont il devient le correspondant, ou avec celle des autres médiateurs, comme celui de la consommation. Nous avons chargé le médiateur territorial de remettre annuellement un rapport d'activité ; ce document peut être source de propositions pour les élus, afin de résoudre des dysfonctionnements aussi bien ponctuels que structurels entre voisins, entre particuliers ou avec l'administration. L'un des apports de cette proposition de loi est d'élaborer un code de déontologie pour tout médiateur territorial en France. Pour cela, elle s'appuie sur des principes inspirés du code de justice administrative, tels que l'indépendance, l'impartialité, la compétence, la diligence et la confidentialité. Afin de garantir, dans la pratique, ces règles déontologiques, le texte prévoit certaines incompatibilités avec des fonctions d'élu ou d'agent territorial de la même collectivité. Ces mesures ont pour objectif d'éviter certains cas, observés notamment lors de mes auditions préalables, de conseillers municipaux de la majorité occupant la fonction de médiateurs territoriaux au sein de leurs communes et statuant sur des litiges survenant avec leur propre administration. d'un amendement de notre rapporteur a permis d'élargir ces conditions d'exercice aux agents contractuels, mais aussi de souligner que la proposition de loi rappelle la gratuité de ce service aux usagers. Enfin, et cela constitue une avancée majeure, cette proposition de loi octroie au processus de médiation territoriale un caractère suspensif. En effet,

Toutefois, si la collectivité pense que la saisie de la médiation n'a que pour seul but de gagner du temps, et si la démarche semble abusive, elle aura le choix de ne pas entrer dans le processus de médiation. De même, si cette dernière n'aboutit pas, le délai de recours reprendra à la date initiale. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, cette proposition de loi ayant pour objet de favoriser le développement des médiateurs territoriaux répond donc à une pratique de résolution de conflits entre l'administration et les administrés. Cette dernière doit être encadrée par la loi, pour ne pas être dénaturée. En rédigeant un nouvel article du code général des collectivités territoriales, ce texte de loi a, je pense, relevé le défi que je lui avais donné avec le sénateur créer un socle de règles communes pour la médiation territoriale, sécuriser son application sur le terrain et faire prospérer ce mode de règlement de conflit de proximité à l'amiable. Voilà ce qui réconcilie la politique et la proximité. Voilà ce qui peut nous réconcilier durablement avec les Français, nous qui nous sommes engagés pour améliorer leur vie quotidienne ». Ce ne sont pas là mes propos,

et même un brin émue de vous présenter ce texte de loi, qui, j'en suis persuadée, répond tant à un besoin de nos collectivités qu'à l'appel lancé par nos concitoyens. La parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

Il tend donc à encourager ce mode alternatif de règlements des litiges, qui nous fait encore trop souvent défaut. La médiation a pour objet principal de prévenir la judiciarisation des litiges. C'est là sa principale vertu. Je vous rappelle sa définition : elle fait intervenir un tiers, le médiateur, qui s'efforce de soumettre aux deux parties une proposition de solution de leur différend, qu'elles sont ensuite libres d'accepter, ou non. Le médiateur, je le rappelle, n'est pas investi du pouvoir d'imposer sa décision, comme l'est, par exemple, le juge. Les collectivités territoriales sont aujourd'hui libres de mettre en place des médiateurs institutionnels pour résoudre à l'amiable les différends pouvant survenir avec leurs administrés.

dans le silence des textes, leurs modalités de nomination et la procédure suivie ne font pas l'objet de garanties légales. De surcroît, leur institution n'est aujourd'hui nullement obligatoire. Le droit en vigueur offre en outre plusieurs autres formes de médiation visant à prévenir la judiciarisation des litiges entre les collectivités territoriales et leurs administrés : je pense au Défenseur des droits, à la médiation administrative, réformée en 2016,

-un travail conjoint, que j'espère fructueux, afin de trouver un accord sur ce texte. Nous sommes convaincus que les collectivités territoriales ont tout intérêt,

Face à ce constat, et reconnaissant l'utilité de la médiation dans les territoires, la commission des lois a souhaité encourager le recours aux médiateurs territoriaux, sans toutefois l'imposer, et ce tout en clarifiant le cadre juridique dans lequel ceux-ci opèrent. Ainsi, nous

Nous avons ensuite renforcé la sécurité juridique du dispositif proposé, sans renoncer à ses objectifs. Pour cela, nous avons mieux défini le champ de compétences du médiateur territorial, en excluant les litiges avec une autre personne publique, de nature contractuelle ou relevant de la gestion des ressources humaines. Nous avons ensuite complété les garanties entourant la nomination et l'exercice des fonctions, en rendant incompatibles les fonctions de médiateur territorial avec celles d'élus ou d'agents des groupements dont serait membre une collectivité territoriale nommant un médiateur. Nous avons aussi clarifié le régime procédural de la médiation territoriale, en faisant de la saisine d'un tel médiateur une cause d'interruption du délai de recours contentieux et en alignant les principes de la médiation sur ceux qui régissent la médiation en matière administrative. Enfin, nous avons adopté des dispositions transitoires pour les médiateurs en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi, et modifié l'intitulé de la proposition de loi, de façon à le mettre en cohérence avec son contenu. Je vous proposerai donc, au nom de la commission des lois, quelques ajustements en séance. Il s'agira notamment de mieux circonscrire les relations contractuelles, que nous souhaitons exclure de la compétence du médiateur territorial. Je vous proposerai qu'il soit incompétent pour traiter des litiges relevant du code de la commande publique, d'une part, et du champ de la médiation de la consommation, de l'autre. En effet, l'un et l'autre font l'objet d'un régime spécifique en application d'une directive européenne, codifiée au titre Ier du livre

De telles pratiques sont bien connues dans le cadre du droit des entreprises. Plusieurs collectivités ont déjà mis en place un médiateur. En effet, sur le fondement des données de l'Association des médiateurs des collectivités territoriales, on peut estimer à environ une cinquantaine le nombre total de médiateurs existants dans les collectivités territoriales et les EPCI. derrière cette proposition de loi est évidemment louable, puisqu'il s'agit de développer et de généraliser de bonnes pratiques, qui permettent parfois de répondre à un besoin de proximité exprimé par nos concitoyens. Pour ce faire, vous avez articulé votre texte autour de deux grands axes. Le premier vise à instituer obligatoirement un médiateur territorial dans les communes de plus de 60 000 habitants et les EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Le second tend à fixer un cadre clair à l'intervention du médiateur territorial

Lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier, le Président de la République a été clair sur la place et le rôle des maires au sein de la République, ainsi que sur sa volonté de faciliter l'exercice de leur mandat.

Pour avoir accompagné le Président de la République lors des 96 heures de débats qu'il a eues avec plus de 5 000 élus locaux, je puis vous dire que le message exprimé par les maires était limpide : « Faites-nous confiance et cessez de nous imposer des normes

Je remercie donc le rapporteur, tout autant que Mme Delattre, d'avoir déposé et fait adopter un amendement en commission tendant à rendre optionnelle, pour toutes les collectivités et leurs groupements, l'instauration de ce médiateur territorial.

en donner quelques exemples. Tout d'abord, qui peut devenir médiateur territorial ? À l'article 1, il est prévu que le médiateur ne puisse exercer une fonction publique élective ou être un agent de la collectivité ou du groupement, ou d'une collectivité appartenant audit groupement.

Et c'est parfois aussi le gage de la proximité, car l'élu connaît la collectivité, mais aussi les citoyens. Ce lien peut être utile dans de petites communes. Il est à noter que le texte prévoit que le médiateur territorial soit le correspondant du Défenseur des droits

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien que la médiation n'ait été introduite dans le code de procédure civile qu'en 1995, elle est une idée très ancienne, profondément ancrée dans l'histoire des relations humaines. Son concept trouve sa racine dans le théâtre grec, où le rôle du médiateur est confié tantôt à un dieu, tantôt à un homme. Aujourd'hui, au sein de nos territoires qui attendent toujours plus de proximité, la médiation démontre bel et bien son utilité et son efficacité comme mode alternatif de règlement des litiges. Au niveau local, un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises par de nombreux maires, désireux de s'inspirer d'une pratique ayant fait ses preuves dans des secteurs très divers. Ainsi, ont été créés des médiateurs municipaux, mais également des médiateurs départementaux et même, plus récemment, un médiateur régional. C'est le cas à Angers, et je salue l'action d'Hervé Carré, qui assure en ce moment même la présidence de la jeune Association des médiateurs des collectivités territoriales. Ces structures de médiation contribuent à rapprocher les usagers de l'administration, en permettant notamment une meilleure compréhension des règles de droit et des pratiques administratives. En outre, elles coexistent avec plusieurs autres formes de médiation, comme le Défenseur des droits ou la médiation administrative. Ainsi, les dizaines de médiateurs, déjà institués dans tous les niveaux de collectivités territoriales, contribuent, par leur action, à éviter complications et conflits juridiques, tant pour les administrés que pour l'administration, ou encore les juridictions administratives, qu'ils peuvent contribuer à désengorger. La proposition de loi que nous examinons cette après-midi vise à conforter cette pratique, en clarifiant les missions du médiateur territorial, en définissant ses obligations et en affirmant son indépendance. Je félicite donc notre collègue Nathalie Delattre d'avoir pris l'initiative de son dépôt. Si je suis je suis profondément convaincu de l'utilité du médiateur territorial, régulateur bienveillant des aléas de la vie administrative, je me félicite également que les travaux sous l'impulsion du rapporteur, aient permis de ne pas accroître inutilement les charges des collectivités territoriales en supprimant le caractère obligatoire de si la consécration législative d'un cadre juridique propre à cette catégorie de médiation apparaît essentielle et nécessaire, il est tout aussi important de laisser les élus apprécier localement et librement leurs besoins, en fonction de leur situation. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité informe d'ailleurs régulièrement les élus de cette possibilité. Ce n'est donc pas l'instrument qui a été remis en cause, mais son caractère obligatoire ; ce dernier a été supprimé à la pleine satisfaction de tous. Je souscris aussi aux modifications apportées par la commission, visant notamment à mieux définir les compétences et les fonctions du médiateur territorial, à garantir son indépendance et son impartialité et, enfin, à mieux encadrer le régime procédural pour assurer sa transparence et sa lisibilité pour les parties. J'ai toutefois déposé deux amendements, afin de ne pas limiter inutilement- à mon sens -et exagérément les missions du médiateur, ce qui ne me semble

elle a fait ses preuves -, il nous apparaît totalement opportun de consacrer dans la loi la possibilité offerte aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'instituer un médiateur territorial.

loi participe à l'enrichissement des débats, afin de faciliter l'exercice des mandats des élus locaux et, au-delà, la vitalité et l'intelligence collective territoriale de l'initiative et de la gestion.

l'ont précisé, la médiation constitue avant tout un mode alternatif de règlement des différends. Elle vise, dans la mesure du possible, à éviter le recours à l'institution judiciaire pour résoudre un conflit. Selon l'Association des médiateurs des collectivités territoriales, il existe déjà une soixantaine de médiateurs dans les différents échelons territoriaux. Cette proposition de loi visait à institutionnaliser le médiateur dans les collectivités locales, avec un seuil minimum pour les communes et les intercommunalités. La commission des lois a souhaité apporter de justes modifications, afin de donner plus de souplesse au dispositif et d'en préciser davantage les contours, en liaison avec l'auteure de la proposition de loi et le pouvoir exécutif. De manière non exhaustive, la commission a rendu facultative pour les collectivités la possibilité d'instituer un médiateur territorial. C'est évidemment une bonne chose le caractère obligatoire nous paraissait également excessif. Elle a ensuite redéfini le champ de compétences du médiateur, en excluant notamment les litiges de nature contractuelle, afin que les litiges relevant de la commande publique ne soient pas concernés. La commission des lois a également souhaité renforcer les garanties entourant la nomination et l'exercice des fonctions, en rendant incompatible celle de médiateur territorial avec celle d'élu ou d'agent des groupements dont serait membre une collectivité territoriale qui nommerait un médiateur. Par souci d'impartialité, nous comprenons parfaitement cette modification. Toutefois, comme le soulignait le ministre Alain Richard en commission, reste en suspens la question de la rémunération au vu de la charge de travail que les fonctions de médiateur peuvent représenter.

Autre clarification apportée par la commission des lois : la saisine du médiateur territorial, qui constitue un motif d'interruption du délai de recours contentieux, sachant qu'elle a précisé que ces nouvelles dispositions ne s'appliqueraient

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois vous dire en préambule que je ne souscris pas à l'exposé des motifs de cette proposition de loi,

Pour ma part, je ne partage pas cette façon de voir les choses, de même que l'hymne au grand débat me laisse quelque peu perplexe. Cela dit, si l'on s'en tient simplement

cette proposition de loi, lorsqu'elle a été présentée à l'examen de la commission des lois, visait à rendre obligatoire la désignation d'un médiateur territorial dans les régions, les départements, les communes de plus de 60 000 habitants et les intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Cette proposition, comme certains collègues l'ont dit, n'est pas nouvelle, puisqu'elle reprend pour l'essentiel un texte de 2014, qu'avaient cosigné, notamment, le président Gérard Larcher et Jacqueline Gourault, aujourd'hui ministre. Mais ce texte n'avait jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat,

s'inscrit aujourd'hui dans un contexte plus favorable, avec à la fois la mise en évidence d'un véritable besoin de médiation et des expériences de plus en plus nombreuses, menées sur une base volontaire. Deux régions, douze départements, vingt-deux communes, deux EPCI : cela commence quand même à être consistant et l'on peut s'en inspirer. Certes, on peut s'interroger sur l'intérêt de la multiplication des textes isolés, qui, par touches fragmentées, abordent la question des relations des citoyens à la collectivité locale, mais ce texte a le mérite de tendre à tirer les enseignements des expériences territoriales qui se sont développées pour donner un cadre juridique unique, avec l'avantage de s'appuyer sur ce qui existe et de créer un socle de règles communes. Par ailleurs, ce texte se distingue de celui de 2014 par le seuil à partir duquel, au départ, il était fait référence, mais aussi par l'intégration des EPCI.

De fait, notre groupe adhère de manière claire à sa philosophie générale, et nous nous sommes appliqués à l'enrichir de manière constructive. Je

nous en étions tous d'accord -, nous souscrivons totalement à la modification adoptée par la commission, sur proposition du rapporteur, tendant à rendre le médiateur facultatif ou optionnel, comme l'a souligné M. le ministre. Deuxièmement, concernant la capacité à être médiateur, nous avons réalisé un travail commun au sein de la commission, pour exclure non seulement les fonctionnaires territoriaux, mais aussi les contractuels, et pour limiter la capacité d'être médiateur à des gens qui n'avaient pas d'intérêt direct à la collectivité ou à la personne morale publique. Nous approuvons aussi les amendements qui tendent à mieux encadrer le cadre d'exercice et les compétences du médiateur, afin d'assurer une plus grande transparence et de la lisibilité pour les parties.

revanche, nous considérons que le texte mérite encore d'être précisé sur les questions de déontologie et d'indépendance du médiateur. Concernant l'incompatibilité du mandat d'élu avec la fonction de médiateur, nous considérions qu'il fallait aller plus loin

dans une société qui se judiciarise de plus en plus et où, malheureusement, les conflits entre les citoyens et l'administration se multiplient, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui privilégie au contraire l'apaisement. Le médiateur territorial est une institution qui existe déjà dans plusieurs communes et qui a fait ses preuves. Il permet de régler les litiges entre les usagers du service public et l'administration territoriale et a donc pour but de créer un climat d'écoute et de compréhension, propice à améliorer la qualité du lien social. Il permet également d'être au plus proche des administrés d'un territoire, et de servir ainsi de correspondant du Défenseur des droits, qui intervient pour les litiges les plus importants. Cette initiative mérite donc un soutien large et transpartisan. Je me réjouis, comme nombre de mes collègues, que le texte de la commission ne fasse de l'instauration de ce médiateur qu'une possibilité et non pas une obligation, comme le texte initial le prévoyait. La souplesse et le cas par cas sont, je crois, comme d'autres matières la clé de la réussite de ce médiateur territorial. Celui-ci doit être au service des collectivités et non pas un énième fardeau pour elles. Vous connaissez le dicton : charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme nous prônons souvent la différenciation territoriale, il eût été incohérent de ne pas appliquer ce principe à cette proposition de loi. Je veux par ailleurs saluer l'initiative de Nathalie Delattre, qui a su être à l'écoute des propositions de la commission des lois. Comme je l'ai dit, ce médiateur existe déjà dans de nombreuses collectivités. Il fallait donc que la loi s'y intéresse, pour le réglementer. Cette proposition de loi est par conséquent bienvenue, puisqu'elle donne une définition du médiateur territorial et précise le régime de cette fonction. La caractéristique première de ce régime est la souplesse dans le processus de désignation, puisque le médiateur peut être désigné par toute personne publique. Il pourra ainsi être installé dans une commune, un département ou encore une région selon les besoins. Néanmoins, le régime se durcit nécessairement s'agissant des incompatibilités et des conditions de son indépendance, et c'est une bonne chose. C'était d'ailleurs une des raisons de la nécessité de légiférer. En effet, il n'est pas tolérable que le médiateur soit une personne qui exerce une fonction publique élective ou qui soit embauchée par une collectivité territoriale ou un groupement. Les dispositions déontologiques contenues dans cette proposition de loi clarifient ainsi son statut, pour éviter toute dérive. Enfin, le rapport que pourra faire ce médiateur territorial permettra d'avoir une meilleure connaissance des points d'achoppement entre les administrés et l'administration. Le médiateur sera également force de proposition, afin de remédier aux problèmes récurrents qui freinent la bonne administration territoriale. En définitive, ce texte a pour objectif de sécuriser juridiquement une fonction qui existe déjà dans certaines dans certaines collectivités et, ainsi, de favoriser un moyen d'apaisement des relations entre les habitants d'une collectivité et leur administration territoriale. C'est également un moyen de désengorger les juridictions.

sans doute parce qu'un bon accord vaut mieux qu'un long et coûteux procès, en 1995, la médiation a été introduite dans le code de procédure civile en France et dans plusieurs autres textes récents sur la résolution amiable des conflits. L'objectif était d'alléger un système judiciaire surchargé et de renforcer les procédures de règlement à l'amiable. La médiation se révèle effectivement utile et efficace

pratiquent quotidiennement l'écoute, la résolution de conflits, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans s'en rendre compte. Une soixantaine de médiateurs a été instituée dans nos collectivités territoriales, principalement dans les communes, alors même qu'aucune obligation Le texte que nous examinons aujourd'hui visait à imposer le recours à la médiation pour régler les litiges pouvant survenir entre les administrés et l'administration publique territoriale et à consacrer juridiquement une nouvelle catégorie de médiateur. Ces objectifs sont louables, et je remercie très sincèrement ses auteurs, sans oublier notre éminent collègue François Pillet, dont l'esprit continue à vivre dans cette maison. Pour autant, tout comme au rapporteur, dont je salue le travail, il nous semblait excessif d'imposer cette nouvelle obligation aux collectivités territoriales. Nous pensons

Le caractère facultatif, que l'auteure de cette proposition de loi a bien volontiers accepté, s'appuiera sur l'esprit de liberté et de responsabilité des élus, qu'il nous faut soutenir, entendre et encourager, comme vous ne cessez de le préconiser, monsieur le ministre, vous qui préférez le sur-mesure à l'uniforme. Toutefois, ce dispositif vertueux mérite toute notre attention. C'est pourquoi nous soutenons les propositions du rapporteur tendant à unifier les règles relatives aux médiateurs territoriaux, à préciser leurs missions, leur périmètre d'action et les critères à remplir pour leurs désignations. seront ainsi principalement chargés de faciliter la résolution des différends entre la collectivité ou l'EPCI et les citoyens. Ils devront exercer leurs fonctions en toute indépendance, ne pouvant recevoir d'instruction de la collectivité. Des règles d'incompatibilité ont également été établies établies pour garantir leur impartialité : le médiateur territorial sera désigné par la collectivité ; un élu ou un fonctionnaire pourra être choisi sous réserve de certaines conditions. Toutefois, Toutefois, la question de la rémunération du médiateur se pose, qui pourrait impliquer mécaniquement un lien de subordination. Comment pourrait-on envisager son indemnisation ? En conclusion, le groupe Union Centriste soutient cette proposition

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner cette proposition de loi visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales, à l'issue des débats menés en amont puis en commission par plusieurs de nos collègues, notamment Nathalie Delattre et François Pillet, qui occupe désormais d'autres fonctions au sein de nos institutions. En découvrant l'intitulé de la proposition de loi, on pense d'emblée aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales au quotidien et que nous cherchons, au Sénat, à réduire ou à résoudre, aux charges supplémentaires, que nous devons prévenir, et aux obligations nouvelles, que nous devons éviter. Toutefois, lorsque l'on examine le texte, on comprend l'intérêt d'une solution qui répond de fait, à un double objectif. proposer, dans la loi, une solution de médiation territoriale, consistant à laisser la possibilité aux collectivités de s'en saisir ou non, tout en harmonisant les pratiques. Cette formule ne doit pas empêcher les collectivités de prévoir d'autres solutions, temporaires ou permanentes, institutionnalisées ou non. Deuxièmement, soutenir et accompagner la mise en oeuvre de procédures alternatives à la saisine du juge, ce que nous appelons les modes alternatifs de résolution des conflits, ou modes amiables de règlement des différends, est aussi une tendance profonde au sein de nos administrations et dans nos sociétés. Mon département, la Vienne, en est un exemple, pour un autre type de médiation, puisqu'il fait partie des départements retenus en 2018 pour l'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire à certains contentieux de la fonction publique territoriale. En instituant un médiateur territorial, on n'institue pas seulement un mode amiable de règlement des différends ; on institue un acteur particulier chargé de répondre à des problèmes ciblés. Cette initiative suscite deux remarques. Premièrement, la priorité doit être celle de la simplification de l'action publique et de nos administrations. À ce titre, l'évolution du texte d'une obligation vers une possibilité offerte aux collectivités territoriales est une bonne chose. Deuxièmement, je relève que le point de vue dominant dans ce texte est celui de l'administration. On peut se poser la question de l'opportunité de consacrer dans la loi une catégorie spécifique de médiateur. La question se pose également du point de vue des usagers : aucune disposition du texte ne leur permet d'identifier les bons services de médiation. Certes, ces médiateurs territoriaux sont considérés, dans la proposition de loi, comme des « correspondants du Défenseur des droits », médiateur plus reconnu par nos concitoyens, mais comment leur permettre de se repérer parmi les différents médiateurs institutionnels, selon la matière visée ? Selon le niveau de collectivité, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, les compétences sont différentes. La question des recours illustre et conforte cette idée d'une complexité accrue pour nos concitoyens., concitoyens., le recours à un médiateur territorial suppose la formation préalable d'un recours gracieux ou hiérarchique. Si nous voulions véritablement Si nous voulions véritablement consacrer cette solution institutionnelle, ne serait-il pas nécessaire, pour simplifier la vie de nos concitoyens et le fonctionnement de nos administrations, de prévoir une suspension des délais de recours contentieux ? Une disposition spécifique dans la loi aurait pu prévoir que la saisine par l'usager d'un médiateur devienne une cause d'interruption du délai de recours contentieux, jusqu'à la fin de la médiation. C'est le cas aujourd'hui dans le cadre des expérimentations de « médiation préalable obligatoire » et pour les organismes de sécurité sociale. il est évident que la médiation ne saurait pallier toutes les imperfections du fonctionnement de nos différents services publics et que le médiateur territorial seul ne saurait permettre à nos administrations d'améliorer leurs fonctionnements et relations avec les usagers. C'est pourquoi, pour terminer sur un point positif, nous devons poursuivre au Parlement, en particulier au Sénat, nos réflexions et travaux en faveur de la simplification de nos services publics et administrations, et au service de nos concitoyens.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, instituer un médiateur territorial dans les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes est incontestablement une bonne chose. chose. Dans une société en proie à de nombreuses tensions, de plus en plus vives, jamais autant qu'aujourd'hui la médiation n'a été à ce point nécessaire. Même s'il ne s'agit pas d'une pratique nouvelle, elle apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. Des médiateurs municipaux ou départementaux ont déjà fait leurs preuves pour régler les litiges entre usagers des services publics et l'administration, mais parfois aussi pour régler des conflits entre habitants et les sempiternelles querelles de voisinage

L'expérience a prouvé que ces institutions se sont révélées efficaces pour prévenir, réduire ou régler des conflits, en créant un climat d'écoute et de compréhension propice à améliorer la qualité du lien social. Résoudre les conflits par le dialogue, restaurer la relation et veiller à ce que les gens se parlent : voilà une très belle ambition à l'heure de l'individualisme forcené et du tout numérique. Recréer du lien social ne devrait pas apparaître comme révolutionnaire. Et pourtant ... En rapprochant les usagers de l'administration, en contribuant à une meilleure compréhension des règles de droit et des pratiques administratives et en proposant des « modifications de comportement », on remet souvent un peu de ce bon sens qui aujourd'hui fait souvent défaut. cela ne peut fonctionner qu'avec un minimum de bonne volonté et de bonne foi, et, surtout, une volonté partagée de sortir de l'impasse : se parler, tout simplement. oui ! Tendre à généraliser cette pratique, oui ; la rendre obligatoire, non ! Je suis donc heureux de constater que la commission a supprimé le caractère obligatoire du recours au médiateur territorial, initialement prévu dans le texte. Là encore, les les collectivités territoriales ont besoin de liberté et de moins de contraintes. Les collectivités territoriales doivent, en fonction de leurs moyens, rester libres de leurs choix, car tout cela a un coût.

Des principes d'indépendance, d'impartialité, de compétence, de diligence et de confidentialité seront réaffirmés dans un code de déontologie. Quant au citoyen qu'un litige oppose à une administration, ses délais de recours seront suspendus le temps de la médiation. Il n'y a donc aucune raison d'aller à l'affrontement. c'est bien volontiers que j'apporte mon soutien à cette proposition de loi, qui a le mérite de remettre une part d'humanité dans un monde administratif parfois considéré comme un monstre à sang froid. Excellent

excessive. En effet, certains des services facturés aux administrés d'une collectivité territoriale ne relèvent pas d'une activité à but lucratif dès lors qu'ils sont en grande partie subventionnés par cette dernière. Songeons par exemple

consommation, en particulier lorsqu'ils mettent en oeuvre un service public industriel et commercial, ou SPIC, qui est légalement considéré comme un service marchand, dès lors que la directive européenne n'exclut pas les « services économiques d'intérêt général » de son champ d'application.

Cet amendement tend à limiter les relations contractuelles qui sont exclues de la compétence du médiateur territorial. Ainsi, le médiateur

a pour objet de rendre incompatibles les fonctions de médiateur territorial avec celles d'agent ou d'élu d'une autre collectivité territoriale membre du même groupement que l'autorité de nomination. Il s'agit d'éviter d'être juge et partie ou d'avoir un intérêt indirect